L’attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023 sur le sol israélien a frappé le monde d’effroi. Plus de 2 000 terroristes islamistes ont assassiné méthodiquement 1 200 personnes et capturé 240 otages. En outre, 40 de nos compatriotes sont morts et 8 sont portés disparus, dont détenus en otage. Dans ce contexte dramatique, la sinueuse stratégie française déroute les Français, comme nos partenaires internationaux. Après avoir rappelé la ligne de la France, le chef de l’État a enchaîné les initiatives controversées. Aujourd’hui, c’est autour d’un éventuel cessez le feu, qui pourrait être mis à profit par les terroristes, que les incompréhensions se cristallisent. Nos diplomates les plus chevronnés expriment des doutes et inquiétudes. Même une certaine presse, qui vous est habituellement favorable, exprime ses graves réserves. Monsieur le ministre, ma question est simple : quelle cohérence dans tout cela ? Quelle initiative d’envergure, concertée et expliquée, la France compte t elle enfin promouvoir pour sortir de cette crise ?

à se défendre légitimement dans le cadre du respect du droit international et du droit humanitaire. Nous avons demandé la libération immédiate et sans condition de l’ensemble des otages. Nous n’avons jamais assimilé le Hamas au peuple palestinien. Nous avons organisé ici même, à Paris, une conférence humanitaire

ministre des armées, est en ce moment même dans les pays du Golfe, pour travailler à cette action diplomatique et éviter une extension du conflit.

à permettre la coexistence du peuple palestinien et de l’État d’Israël. Cette solution à deux États est la seule qui permette à ces deux peuples de vivre en paix et en sécurité, l’un à côté de l’autre. La Monsieur le ministre, la diplomatie gaullienne, c’est être capable de parler à tout le monde et non dire à chacun ce qu’il a envie d’entendre.

Dernièrement, les relations se sont tendues avec les Israéliens, en raison de déclarations ambiguës du chef de l’État. Quant aux pays arabes, ils n’ont fait que nous recevoir poliment. Selon moi, ce n’est pas notre outil diplomatique qui est en cause, mais le pilotage politique au plus haut niveau.

Cet accord est d’une importance majeure pour nos concitoyens, mais aussi pour nos entreprises et nos collectivités. En effet, EDF s’y engage à vendre son électricité nucléaire à un prix évalué à 70 euros le mégawattheure en moyenne. Après un an de négociations intenses et après avoir obtenu gain de cause au niveau européen sur la décorrélation du coût de l’électricité de celui des énergies fossiles, notamment du gaz, la France reprend enfin le contrôle sur les prix de l’électricité. De plus, alors que la régulation actuelle ne portait que sur un tiers de la production, ce nouvel accord concerne l’intégralité de l’électricité produite, ce qui permet à EDF de gagner en visibilité, facteur essentiel pour un acteur industriel, comme pour nos concitoyens et nos collectivités.

force est de constater que nous devons apporter des précisions aux consommateurs. Ainsi, monsieur le ministre, quel sera l’impact de cet accord sur la facture de nos concitoyens et des entreprises en 2025 ?

cet accord garantit la compétitivité de nos entreprises industrielles grâce à l’un des prix les plus compétitifs de tous les pays européens. C’était notre priorité absolue. En deuxième lieu, il garantit la stabilité aux ménages – c’était notre deuxième priorité. Il n’y aura pas de ressaut entre fin 2025 et début 2026, puisque les prix seront étalés dans le temps. Nous ne voulons pas que les ménages connaissent de nouveau une explosion des prix comme celle qu’ils ont connue pendant la crise énergétique. Enfin, en troisième lieu, cet accord garantit la rentabilité d’EDF : ce n’est pas parce qu’elle est à 100 % publique qu’EDF doit

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France entière est traumatisée par la multiplication des actes antisémites dans notre pays. Ceux ci appellent une condamnation unanime.

Nous ne devons pas tolérer le cancer de la haine au sein de notre nation. Ce cancer n’est, hélas !, pas nouveau. Nous le pensions en rémission, mais les événements au Proche Orient le mois dernier ont entraîné une forte résurgence de ces actes. Monsieur le ministre, pouvez vous nous donner le bilan exact de ces agressions ? Combien ont fait l’objet de poursuites et de condamnations ? Les Français ont besoin de savoir ; ils attendent de la fermeté dans la réponse judiciaire. Parallèlement, par des incitations à la haine relayées sur les réseaux sociaux, des puissances étrangères tentent de déstabiliser notre pays. L’affaire des couples moldaves peignant des étoiles de David sur des immeubles en est la dernière illustration.

La désinformation et les manœuvres de la cyberguerre sont en train de tuer la démocratie. Nous en sommes depuis longtemps déjà la cible, tant à l’étranger que sur notre propre sol. Il nous faut répondre. Comment le Gouvernement lutte t il contre les tentatives étrangères de désinformation ? La parole

dans les 950 lieux que les Français de confession juive fréquentent, notamment les écoles ou les synagogues. Ces événements ont donné lieu à 571 interpellations, dont 130 d’étrangers.

Les deux couples ont quitté le territoire national. Le premier a été interpellé et expulsé, après des interrogatoires. Des éléments extrêmement précis nous amènent à penser qu’un commanditaire étranger a une part de responsabilité dans cette situation.

Vous avez tenté de les rassurer tant sur leurs moyens que sur leur avenir institutionnel, troublé par la nouvelle mission Woerth. Force est de le constater, l’effort consenti par votre gouvernement ne répond pas totalement aux besoins exprimés par les départements,

Vous avez rappelé le rôle indispensable des départements. Il s’agit aujourd’hui de les soutenir, pour maintenir,, la démocratie locale et leurs investissements.

Fraîchement élu dans le Lot et Garonne et ancien vice président du département, je demeure attaché à cette collectivité de proximité, qui supplée les services de l’État, notamment dans les zones rurales. Madame la ministre, comptez vous intégrer aux projets de loi d’examen des mesures plus que significatives pour permettre aux départements de retrouver leur autonomie financière et d’assurer sereinement leurs missions de solidarité

qu’il avait le souci de maintenir cette proximité et de la recréer là où elle n’existe pas suffisamment ou bien là où elle n’existe plus. Sur bien des sujets – aménagement du territoire, politique sociale, transition écologique et service public –, la maille départementale est une maille pertinente, pertinente, qui permet de travailler à l’échelle d’un territoire cohérent tout en conservant une capacité d’action de proximité à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Notre réflexion se fera donc à l’aune du rôle essentiel des départements dans l’actuelle organisation territoriale. J’en suis convaincue, tout comme l’est la Première ministre,

a débloqué en faveur des départements : 150 millions d’euros pour l’autonomie, 100 millions d’euros pour répondre à la problématique des mineurs non accompagnés et 100 millions d’euros pour les départements en situation de fragilité. Oui, monsieur le sénateur, nous veillons sur nos départements. La parole le savez, madame la ministre, les départements sont des collectivités essentielles pour l’équilibre de nos territoires. Premiers financeurs de la solidarité, premiers aménageurs, ils sont aujourd’hui les acteurs publics locaux reconnus de l’égalité et du maintien des services publics. Rétablir l’autonomie financière des départements est un enjeu qui dépasse le seul échelon départemental. J’espère votre soutien plein et entier au maintien des départements au sein de l’architecture territoriale, afin de « figer » les territoires actuels.

Monsieur le président, madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous examinons cette semaine le budget de la sécurité sociale. Le Gouvernement

Une telle trajectoire est totalement inédite, alors même que la crise sanitaire et ses effets sont derrière nous. Ma question est très simple : pourquoi n’êtes vous pas capables de remettre les finances sociales à l’équilibre ? Avez vous baissé les bras ? Avez vous renoncé ? La parole est à M. le ministre de la santé et de la prévention. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bernard Jomier, le Gouvernement présente en effet un projet de loi de financement de la sécurité sociale visant à ramener le déficit de la branche maladie, qui était de 22 milliards l’an dernier, à 8,8 milliards d’euros, sur un total de 255 milliards d’euros de dépenses.

! On pourrait accepter des déficits si l’hôpital allait mieux qu’il y a cinq ou six ans, mais l’hôpital se dégrade, les personnels s’en vont et l’offre de soins se contracte. On pourrait accepter des déficits si nos concitoyens, sur tout le territoire, avaient accès aux soins de proximité et à un médecin généraliste, mais les déserts médicaux se répandent et les pénuries s’accroissent. Vous êtes donc en échec : ce sont des vagues de mauvais résultats dans un océan de déficit. Monsieur le ministre, votre gouvernement gère mal la sécurité sociale. La parole est à Mme Cathy Apourceau Poly, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste Monsieur le ministre, le Pas de Calais connaît depuis deux semaines les inondations les plus catastrophiques du siècle. Plus d’un tiers des communes sont touchées : habitations, entreprises, exploitations agricoles ou bâtiments publics.

Ils souhaitent une simplification des procédures qui leur permettrait d’intervenir, entre autres, en matière d’entretien des marais et des fossés. Merci à tous ces volontaires – anonymes, associations, pompiers, sécurité civile, agents communaux et services de l’État – qui font un travail admirable. la visite du Président de la République nous a donné l’espoir d’une implication durable de l’État. Les premiers actes attendus par la population pour résoudre les problèmes ont été posés. Les 50 millions d’euros d’aide d’urgence sont un premier pas. Toutefois, à l’évidence, nonobstant la participation des assurances, les investissements nécessaires pour reconstruire, puis prévenir de telles catastrophes, feront exploser cette enveloppe.

des entreprises partiront, des agriculteurs jetteront l’éponge et la désespérance s’ancrera dans la population. Pouvez vous, monsieur le ministre, nous éclairer sur la réflexion de l’État et la réponse qu’il entend apporter aux propositions du président de la région des Hauts de France et du président du département du Pas de Calais ? La parole

Les attentes sont de tous ordres : financier, juridique opérationnel. Financièrement, d’abord, il est impossible aujourd’hui d’avancer un chiffrage des dégâts et des désordres pour les habitants, mais également pour les commerçants, artisans, agriculteurs, entrepreneurs. Quoi qu’il en soit, il est à présent indispensable de simplifier et d’accélérer les procédures administratives pour permettre à chacun de reprendre une vie normale. Juridiquement, ensuite,

essentiellement de conditions environnementales excessives. Monsieur le ministre, avec le réchauffement climatique, ce type d’événements risque de se multiplier. Les séquelles sont matérielles, mais également psychologiques. Il faut conclure !

dernière. Aujourd’hui même, une proposition de simplification sur les curages des rivières a été transmise au Conseil d’État. Ce sujet ne concerne pas que le Nord et les Hauts de France

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, demain, jeudi 16 novembre, les États membres de l’Union européenne sont appelés à voter sur la réautorisation pour dix ans du glyphosate. dans lequel la France aura un rôle déterminant, a une importance cruciale, alors que les preuves s’accumulent sur les dangers de cette molécule pour la santé et l’environnement. Vous le savez, le glyphosate est classé comme cancérogène probable depuis 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer

Si la France s’abstient de nouveau, demain, sur le glyphosate, elle portera une lourde responsabilité. Pourtant, on s’en souvient, le Président de la République annonçait en 2017 une sortie de son usage en France sous trois ans, souhaitant entraîner l’Europe entière derrière lui. Aujourd’hui, on constate un abandon de tout leadership sur la question. La France a quitté le wagon de tête pour être en queue de train, avec un discours à géométrie variable. Un jour, le prétexte national pour l’inaction est la distorsion de concurrence avec nos voisins. Aujourd’hui, vous ne montrez aucune ambition à l’échelle européenne, alors que d’autres États membres ont pris des positions bien plus courageuses. Monsieur le ministre, la France votera t elle contre la réautorisation du glyphosate ? Êtes vous prêt à jouer votre rôle pour son interdiction rapide au niveau européen ?

La position de la France est simple : partout où l’on peut réduire les usages, conformément à la trajectoire que nous nous sommes donnée, nous le faisons ; et là où il y a des impasses, nous assumons aussi les positions qui sont les nôtres. Nous continuerons donc à défendre au niveau européen la volonté de réduire l’usage du glyphosate

Monsieur le ministre, vous le savez parfaitement, la fabrique du doute fonctionne à plein régime aujourd’hui avec des pseudo études scientifiques payées par les grands groupes.

Ne la gâchez pas, ne faites pas en sorte que nous ayons honte de la position de notre pays ! Le glyphosate, c’est chose avérée, est un poison : des méta analyses le prouvent tous les jours et ce ne sont pas de petites études faites par les grands groupes

Le rouge et l’orange : ces deux couleurs sont désormais familières, mais si angoissantes pour les habitants du Pas de Calais. Mes premiers mots iront donc vers les sinistrés des deux tempêtes et des inondations, qui se prolongent depuis trois semaines.

Je pense aux sinistrés agricoles, qui n’ont plus de champ à semer, plus de bêtes à faire pâturer, plus de légumes à récolter. Je pense aux sinistrés économiques, qui ne peuvent plus faire fonctionner leurs entreprises ni faire travailler leurs salariés. Jamais nous n’avons connu de catastrophe d’une telle ampleur, avec une étendue géographique si importante. Jamais nous n’avons autant souhaité la solidarité locale et nationale pour venir effacer le désespoir d’un avenir sombre, encore à découvrir. Au delà de la solidarité des collectivités locales, déjà précisée et qui va s’accroître, au delà de la solidarité nationale, pleinement assurée dans l’urgence par nos préfets et leurs services, la représentation nationale et les collectivités attendent des précisions pour le futur de ces sinistrés. Nous avons aussi besoin d’une solidarité européenne. Comme je l’ai rappelé au Président de la République hier, je souhaite que l’on puisse d’ores et déjà activer les trois mécanismes de soutien européen

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, oui, nous avons activé les dispositifs européens. Nous allons même un peu plus loin,

plutôt que de dépenser trop d’argent en études incessantes, usantes, traînantes et parfois inutiles ! La parole est à Mme Corinne Féret, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

dilemmes éthiques intenables » auxquels ils sont confrontés, faute de lits et de personnels dans nos hôpitaux. Partout, dans mon département du Calvados comme ailleurs, les soignants alertent sur la dégradation sans fin de leurs conditions de travail. Ils indiquent ne pas avoir choisi de travailler à l’hôpital pour être contraints de trier les patients ou d’être maltraitants. Voilà quelques mois, le service statistique du ministère de la santé indiquait que plus de 21 000 lits avaient été supprimés entre 2017 et fin 2021, soit l’essentiel du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Dans 163 villes de France, les urgences ont été ponctuellement fermées cet été

Pas une semaine ne passe sans que l’état de délabrement des secteurs de la psychiatrie ou de la pédiatrie, abandonnés de l’État, fasse la une, sans parler de toutes ces maternités que vous avez laissées se dégrader au point que plus personne ne veuille y travailler. Monsieur le ministre, il faut sortir des logiques comptables technocratiques ! Allez vous enfin écouter les professionnels de terrain, garantir un nombre maximal de patients par soignant, comme le Sénat l’a voté, et donner à l’hôpital public les moyens de prendre correctement en charge les patients ?

l’hôpital public, est dans une situation difficile. Il connaît une crise dont les racines sont profondes et qui fait écho, en partie, à la question de votre collègue Bernard Jomier voilà quelques L’avantage d’avoir un peu d’expérience, c’est de pouvoir revenir sur certaines de ses propres erreurs. En 2017, la sécurité sociale et la branche maladie étaient à l’équilibre, en effet, mais sans doute l’hôpital avait il été la variable d’ajustement de ces dépenses. Nous étions peut être allés trop loin dans la régulation financière à cette époque.

Nos hôpitaux doivent demeurer des lieux de soins sûrs et humains. Les Français comme les soignants attendent des actes forts ! La parole est à M. Laurent Duplomb, pour le groupe Les Républicains. alimentaire. Monsieur le ministre, il y a aujourd’hui deux types d’acteurs : ceux qui veulent une agriculture qui rime avec environnement et qui croient au progrès, et ceux qui considèrent que l’agriculture s’oppose, par nature, à l’environnement et veulent l’éradiquer.

qui partaient pourtant d’un bon principe, le Parlement européen veut désormais interdire toute pratique, sauf en agriculture biologique, secteur pourtant en crise de surproduction.En résumé, soit les agriculteurs se convertissent et vendent à perte, soit ils s’arrêtent tout de suite ! C’est faux ! Autrement dit, pour protéger ces zones, comme je l’avais déjà souligné voilà deux ans ici même, on accepte de rayer l’agriculture de la carte. En France, Natura 2000, c’est 7 millions d’hectares, dont près de 5 % de la surface en production fruitière et 70 000 hectares de grandes cultures pour la seule Beauce. Après le, cette nouvelle décision décroissante de gens qui préfèrent une agriculture importée est contraire à notre souveraineté, dont votre ministère porte le nom. en préambule, il y a deux camps : ceux qui croient en une agriculture de progrès et ceux qui veulent éliminer l’agriculture. Je fais partie du premier camp et je m’opposerai à ce projet de décision européenne. Monsieur le ministre, dans quel camp êtes vous ? La parole est à M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs,

Monsieur le ministre, qui voulons nous protéger ? Toutes les trois minutes, un enfant est victime de violences sexuelles. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Au total, 5 millions d’adultes ont subi des violences sexuelles dans leur enfance.

En 2021, le Président de la République a promis à toutes les victimes qu’elles ne seraient plus jamais seules. En 2021, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences faites aux enfants a été créée pour une durée de trois ans. Ses travaux doivent s’achever le 31 décembre La Ciivise est devenue un espace reconstructeur, qui accompagne les victimes. Se pose donc la question de son maintien. En trois ans, elle a accompli un travail titanesque et salvateur. Elle a recueilli recueilli près de 30 000 témoignages. En trois ans, la Commission a fait des propositions fortes avec pour seule boussole la volonté de protéger enfin les mineurs et de condamner les agresseurs.

nous en savons quelque chose au Sénat. Le juge Édouard Durand, avec son expertise, sa détermination, ses convictions, a démontré qu’il était l’homme de la situation. La Ciivise ne peut se passer du juge Édouard Durand

quelles réformes structurantes et puissantes allez vous proposer pour répondre, non pas à une crise, mais plutôt à un échec majeur de notre système éducatif

j’ai eu l’occasion de le dire dès ma nomination au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, mon objectif est l’élévation du niveau général de nos élèves. Tous les chantiers que j’ai ouverts doivent y concourir. Quand on travaille pour restaurer l’attractivité du métier d’enseignant, on agit pour élever le niveau de nos élèves. Quand on travaille pour restaurer l’autorité du maître à l’école, on agit pour l’élévation du niveau des élèves. Quand on réforme le lycée professionnel, Carole Grandjean et moi même le faisons, on agit pour l’élévation du niveau

Songez qu’un élève sur quatre, à l’entrée en quatrième, n’a pas le niveau de lecture attendu en fin de CM2 ! Eh oui ! Je présenterai, au début du mois de décembre, des mesures fortes pour l’élévation du niveau général à l’école et au collège. Je le dis : je n’ai aucun tabou.

En 2018, le Président de la République avait annoncé vouloir « répondre aux défis du vieillissement ». La proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France sera examinée la semaine prochaine à l’Assemblée nationale. Une enquête récente, menée par la Fédération hospitalière de France, a révélé que 85 % des Ehpad se trouvaient en situation déficitaire à la fin de l’année 2022. Ces déficits tendent à devenir structurels et croissants dans ce secteur – pour ne pas dire, hélas !, qu’ils le sont déjà. J’ai été alerté, hier, sur la situation budgétaire de plusieurs Ehpad de mon département.

faites vous le choix de délaisser nos aînés ? Faites vous le choix de délaisser le personnel des Ehpad, qui travaille dans des conditions déjà très difficiles ? L’État doit être à la hauteur de ces enjeux. Je suis persuadé que l’ensemble de mes collègues ici présents sont d’accord avec moi. moi. Dès lors, ma question est simple et appelle une réponse concrète : le Gouvernement envisage t il de mettre en œuvre des compensations financières pérennes et intégrales ?

œuvre des politiques publiques beaucoup plus lisibles et augmenter ainsi la prise en charge par l’État. Ce que nous avons mis sur la table, et je crois que les départements sont en accord avec cette proposition, c’est que 50 % de

Monsieur le ministre, le 8 novembre dernier, par la voix de sa présidente, Mme von der Leyen, la Commission européenne a recommandé officiellement l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Ukraine. Cet avis favorable doit être approuvé à l’unanimité par les Vingt Sept lors du prochain Conseil européen des 14 et 15 décembre prochains, Sans évoquer la question diplomatique que pose cette initiative, dans un contexte de recherche de paix et de désamorçage du conflit, je souhaite vous poser la question fondamentale de la préservation de nos intérêts agricoles. Vous revenez d’Ukraine, où vous avez annoncé œuvrer au « renforcement de la coopération agricole entre nos deux pays » et travailler avec cet État sur le chemin de son adhésion à l’Union européenne et invoqué la « solidarité » des agriculteurs dans le contexte de « l’ouverture du marché européen aux produits agricoles ukrainiens ». Monsieur le ministre, pourriez vous nous éclairer sur vos intentions ? Si la position favorable de la France ne fait désormais aucun doute, êtes vous bien conscient du désarroi des agriculteurs français, pris en étau entre des normes européennes toujours plus exigeantes et complexes, une ouverture toujours plus grande à la concurrence, avec la multiplication des accords de libre échange, et une envolée du coût des intrants et de l’énergie ? Monsieur le ministre, quels intérêts défendez vous ? Votre dernière déclaration, largement relayée par vos soins sur les réseaux sociaux, sonne comme une volte face pour de nombreux syndicats agricoles. Nous ne pouvons prendre le risque de sacrifier nos intérêts. Comment allez vous protéger l’agriculture française dans une telle perspective ?

Il est vraiment temps de défendre avec force l’agriculture française. Notre souveraineté alimentaire doit être une vraie priorité nationale ! La parole est à M. Bruno Rojouan, pour le groupe Les Républicains.

En effet, sommés de se mettre aux normes dans des délais intenables, les petits propriétaires bailleurs concernés par les rénovations thermiques – ils sont nombreux en France – font leurs comptes. Or, en termes d’équilibre financier, Si, pour les secteurs géographiques des métropoles, où les loyers sont plutôt élevés, on peut tendre vers un équilibre sur un nombre d’années acceptable, ce n’est absolument pas le cas

les charges des travaux des revenus locatifs, est doublé jusqu’en janvier 2025 pour des travaux permettant d’atteindre la performance de classe D. Si j’ajoute à cela le

inégalé : la construction de logements neufs est bloquée ; l’achat vente de logements anciens est au plus bas depuis des décennies ; et là,

est reprise. Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ayant été transmis au Sénat, le groupe de travail dont les membres ont été nommés en séance le 8 novembre dernier peut être transformé en commission spéciale. Il n’y a pas d’opposition ? Il en est ainsi décidé. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est parvenue à l’adoption d’un texte L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2024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

Selon l’Insee, au cours du premier semestre 2021, le taux de marge des entreprises atteignait près de 36 %, un niveau jamais atteint depuis 1949. Parallèlement, l’Institut de recherches économiques et sociales évalue le montant des aides publiques reçues par les entreprises à 8,4 % du PIB, ce qui en fait l’un des plus hauts de l’OCDE. Dans ce contexte, il nous semble important de limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonération de cotisations sociales. que tout nouveau dispositif d’exonération soit compensé par la suppression d’une exonération existante pour un montant équivalent, afin de ne pas affaiblir la sécurité sociale. La

de compensation systématique et intégrale de toute nouvelle exonération de cotisations sociales, par la suppression, dans le même temps et dans les mêmes proportions, d’un dispositif d’exonération existant pour un montant équivalent. Le coût total des mesures d’exonération prétendument en faveur de l’emploi a atteint 73,8 milliards d’euros en 2021 pour l’ensemble des régimes de sécurité sociale,

selon lequel toute mesure d’exonération générale de cotisations à la sécurité sociale devrait systématiquement être compensée par l’État. Cela n’est plus le cas, loin de là ! On assiste à de nombreuses exonérations. Vous en inventez très régulièrement de nouvelles,

est à Mme Nadège Havet. Pour contribuer au développement de l’usage du vélo pour se rendre au travail, une participation obligatoire de l’employeur, à hauteur de 50 % des frais de location de vélos engagés par les employés, existe déjà, au même titre que

Le transport public étant la colonne vertébrale d’une mobilité durable, il faut permettre aux employeurs de participer davantage à la prise en charge des abonnements de transport public de leurs employés. Jusqu’à l’été 2022, la loi prévoyait certes une exonération de cotisations et de contributions sociales,

Le Gouvernement ayant pérennisé ce dispositif pour l’ensemble des fonctionnaires depuis le 1 septembre dernier, il serait juste que les salariés du secteur privé puissent continuer d’en bénéficier au delà de 2023. Ainsi, sur la base du volontariat

à l’employeur de prendre en charge une fraction supérieure à 50 % du coût des titres d’abonnement, voire la totalité. Dans ce cas, la participation facultative – au delà de 50 % – est exonérée, dans la limite des frais réellement engagés, soit jusqu’à 100 %.

particulièrement dans les secteurs fruitiers et les vendanges. Notre économie touristique repose également sur ces travailleurs indispensables à nos entreprises. Ceux ci souffrent néanmoins d’une situation particulièrement précaire, ce qui rend ces métiers peu attractifs discontinuité des revenus, faible protection sociale, difficultés de l’accès au logement. Ainsi observe t on une pénurie de main d’œuvre qualifiée, récurrente dans ce domaine, qui oblige de nombreux employeurs à recourir à des travailleurs étrangers, voire illégaux. Il est donc nécessaire de favoriser le recrutement par des mesures fiscales incitatives, afin de répondre aux difficultés de logement des saisonniers dans les zones touristiques et agricoles. À cette fin, le présent amendement tend à exclure de l’assiette des cotisations et de la CSG les avantages en nature que représentent les logements des saisonniers, pour une durée n’excédant pas six mois. Quel

le rétablissement des cotisations patronales à la branche maladie. Vous le savez, depuis 2015, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a permis d’exonérer les employeurs de 6 points de cotisations sociales, et sa transformation en réduction pérenne des cotisations maladie pour les employeurs n’a eu aucun effet, ou si peu, sur la création d’emplois en France. Pis, cela a contribué à aggraver la situation des comptes sociaux, avec une perte de recettes pour l’État et la sécurité sociale d’un montant de 28 milliards d’euros pour 2024. Au travers de cet amendement, nous proposons une

des ménages. La sécurité sociale rembourse 92,8 % des soins hospitaliers et 92 % des transports sanitaires, contre seulement 69,2 des soins de ville, 73,8 % des médicaments et 45 % des autres biens médicaux. Le montant total des dépenses d’un remboursement intégral par l’assurance maladie peut être estimé autour de 24,5 milliards d’euros. Ce montant serait largement inférieur si l’on tenait compte des effets directs ou indirects d’un remboursement à 100 %. Cela n’entraînerait évidemment pas la suppression des complémentaires santé. Le ministre de la santé a indiqué vouloir opérer un virage en termes de prévention ; il nous semble que ces organismes pourraient y contribuer. Quel

à l’exclusion de la fiscalité, comme la TVA, par exemple. Cet amendement est le reflet de la vision à la fois traditionnelle et cohérente du groupe CRCE K, qui repose sur un financement assurantiel de la sécurité sociale, c’est à dire par des cotisations et des recettes assimilées. assimilées. Je rappelle qu’historiquement l’apparition puis l’augmentation de la fiscalisation des recettes de la sécurité sociale sont liées à la CSG et que l’instauration de cet impôt est une réponse des pouvoirs publics à des déficits déjà récurrents. On ne peut donc opposer un « âge d’or » de la cotisation à la misère du financement mixte. Par ailleurs, la majorité sénatoriale assume, d’une part, les choix opérés par le passé pour limiter l’écart du coût du travail entre la France et ses concurrents et, d’autre part, le choix de compenser les pertes qui en résultent pour la sécurité sociale, et donc le caractère mixte.

monsieur le ministre,

Contrairement aux CIAS, les EPCI ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile. Le Gouvernement avait en effet indiqué vouloir réserver l’exonération aux structures spécialisées. Nous proposons donc une exonération pour les EPCI ayant pour objet l’action sociale. Quel

D’après le dernier rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS), la croissance des allégements généraux de cotisations a été encore plus soutenue en 2023, à hauteur de 12 %.

pointé du doigt les effets de seuil du dispositif Fillon. Ces critiques sont alimentées par le phénomène de tassement de la distribution des salaires actuellement observable en France. En effet, 50 % des salariés gagnaient moins de 2012 euros net par mois en 2021, soit environ l’équivalent de 1,6 Smic.

en 2022. Du point de vue macroéconomique, ces données semblent donc accréditer l’hypothèse de l’existence de trappes à bas salaires. Nous proposons par conséquent de revenir sur ce dispositif, qui entraîne par ailleurs une remise en cause du pacte social.

Nous proposons ainsi de conditionner les exonérations dites Fillon au développement de l’emploi, à la revalorisation des salaires, aux engagements qui visent à favoriser l’investissement à la prise en compte des critères environnementaux. L’arrêt des exonérations de cotisations et la fin des niches fiscales sont les éléments essentiels d’une croissance de l’emploi, des salaires et du financement de la sécurité sociale. Il s’agit simplement de conditionner ces 26 milliards d’euros. L’amendement n°

vous. Au contraire, je vous invite à combattre pour nos droits. Et vous, messieurs, chers collègues, je vous appelle à faire de même. Les femmes gagnent en moyenne encore 25 % de moins que les hommes.

leurs obligations en matière d’égalité salariale. Quoi de plus simple ? d’un accord relatif à l’égalité professionnelle. La France est en effet à la quinzième place du classement du Forum économique mondial sur l’égalité professionnelle. Monsieur le ministre, soit vous nous accusez de vouloir infliger un choc fiscal à notre pays,

Il y va également de l’équité de traitement entre les employeurs de la fonction publique et du respect du principe d’égalité entre les agents publics. Quel est l’avis de la commission ? La commission et le Sénat

d’un contrat collectif obligatoire, qui constitue objectivement la formule permettant la plus grande mutualisation des risques sur une base solidaire. Il paraît donc opportun de réserver les avantages fiscaux et sociaux liés à ces cotisations à des assurances souscrites

mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinction entre les périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. On observe également une raréfaction de la commande des bailleurs sociaux, en proie, notamment, à un manque de foncier, alors demande croissante. La réorientation annoncée du prêt à taux zéro et le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du dispositif achèvent de perturber le secteur. Et je ne parle pas de la flambée des prix des matériaux de construction, des surcoûts liés à l’augmentation des délais d’approvisionnement ni du contexte spécifique du bâti tropical, qui ont une incidence locale considérable sur le coût de construction. Or l’intégralité des surcoûts est pour l’heure à la charge des seules entreprises du secteur du BTP, alors que celles ci sont, comme la majeure partie des entreprises ultramarines, confrontées

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur.

surcoûts liés à l’augmentation des délais d’approvisionnement ni du contexte spécifique du bâti tropical, qui ont une incidence locale considérable sur le coût de construction.

un certain nombre de dispositifs : le gel des pénalités de retard des entreprises du bâtiment, la mise en place d’une médiation de filière pour le BTP, la réactivation des cellules de crise ou encore une aide temporaire consistant

pour cet amendement, c’est apporter notre soutien à ce secteur, qui connaît des difficultés de recrutement et qui doit parfois faire face à des conditions climatiques difficiles. Adoptons cette mesure qui permettra de donner un peu de quiétude et d’espérance à notre ruralité.

Certes, l’article 20 du projet de loi de programmation des finances publiques prévoit que les niches sociales instaurées par un texte promulgué à compter du 1 janvier 2023 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois

aux lois de financement de la sécurité sociale impose l’évaluation systématique de tous les dispositifs d’exonération. Il serait paradoxal de plaider pour des évaluations régulières des exonérations et des niches tout en pérennisant un dispositif d’exonération

Le dispositif TO DE représente un soutien vital pour les agriculteurs employeurs de main d’œuvre. Néanmoins, certains employeurs agricoles ne peuvent bénéficier de ces exonérations. C’est notamment le cas des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (Etarf), alors qu’elles sont confrontées à une augmentation importante de leurs coûts d’exploitation. En effet, depuis la loi de finances pour 2015, ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif et aux travaux forestiers, « à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers Pourtant, ces entreprises, qui emploient 15 % des salariés de la production agricole, sont confrontées, comme les autres, à une perte de compétitivité, la crise sociale, économique et maintenant énergétique n’ayant pas arrangé les choses. C’est pourquoi nous proposons que les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers puissent bénéficier

Nathalie Delattre. Cet amendement vise à améliorer le dispositif spécifique d’exonération de cotisations et de contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole, en faisant passer le seuil de dégressivité dégressivité de 1,2 à 1,25 Smic. Nos filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture sont confrontées au dumping social de nos concurrents européens, notamment de l’Espagne, de l’Italie ou de l’Allemagne,

Nous proposons donc d’augmenter le seuil de dégressivité, afin de mieux prendre en compte la réalité des rémunérations des salariés agricoles concernés, en particulier en cette période d’inflation. Quel

En effet, à ce jour, seules les exploitations agricoles bénéficient de l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi. Or les coopératives de fruits et légumes sont dirigées par les exploitants agricoles produisant les fruits et légumes des employeurs agricoles. Elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. À ce titre, et selon la même saisonnalité que leurs adhérents, les coopératives qui conditionnent des fruits et légumes sont amenées à embaucher un grand nombre de saisonniers. Or leur exclusion du bénéfice du TO DE freine ces embauches, ce qui pénalise le développement de l’emploi en agriculture, pourtant un élément important de la compétitivité de la ferme France.

visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a instauré, sur l’initiative du Sénat, un dispositif de réduction de cotisations patronales en contrepartie de la mise à disposition

Le bénéfice de cette réduction de cotisations patronales pour les employeurs publics paraissait pourtant parfaitement justifié, pour les communes rurales, pour lesquelles la mise à disposition de leurs employés constitue une charge non négligeable. En excluant les employeurs publics du dispositif, le législateur s’est donc privé, dans un contexte de crise du volontariat, d’un vivier de recrutement de sapeurs pompiers volontaires significatif, alors même que la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France (FNSPF) s’est donné pour objectif de recruter 50 000 volontaires d’ici à 2027 pour répondre à l’augmentation de la sollicitation opérationnelle à laquelle sont confrontés les Sdis. Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en modifiant l’article 52 de la loi du 10 juillet 2023 de manière à inclure les employeurs publics dans le champ des bénéficiaires potentiels du mécanisme de réduction des cotisations patronales accordé en contrepartie – j’y insiste – de la mise à disposition de leurs employés sapeurs pompiers volontaires au profit des Sdis. Quel

La volonté des rapporteurs était non pas de réduire la portée du dispositif en introduisant cette limitation de temps, mais uniquement de garantir sa recevabilité au regard du domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

Il est en effet essentiel que le mécanisme de réduction de cotisations patronales accordée en contrepartie de la mise à disposition par les employeurs de leurs salariés sapeurs pompiers volontaires s’inscrive dans le temps long afin de maximiser la portée incitative du dispositif dans un contexte de crise – je me permets d’insister – du volontariat des sapeurs pompiers. Le présent amendement vise donc à pérenniser la mesure, conformément à la volonté initiale des auteurs de la proposition de loi. Quel

société de confiance, dite loi Essoc, cet amendement vise à créer les conditions pour faciliter le recours au relayage sur le temps long afin d’apporter durablement une solution de répit adaptée aux proches aidants.

L’établissement public national Antoine Koenigswarter accompagne, dans une grande majorité de régions de métropole et d’outre mer, plus de 5 000 personnes de tous âges en situation de handicap dans le cadre d’environ quatre vingts unités. L’article 23 de la loi du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social fait obligation à l’Epnak

bénéficié du dispositif de réduction progressive des cotisations sociales employeur dès son entrée en vigueur dans les années 2000 et pendant plusieurs années, avant d’en être privé par des décisions de l’Urssaf d’Île de France en 2019 puis en 2021, validées par un jugement du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire d’Évry. La non éligibilité au dispositif d’exonération des cotisations employeur a pour effet de provoquer un surcoût sur la masse salariale de l’établissement et d’entraîner une distorsion avec d’autres structures médico sociales. Le présent amendement a donc pour objet de permettre à l’Epnak de bénéficier de nouveau, à compter de 2024, du dispositif de réduction progressive des cotisations sociales employeur.

l’expérimentation, qui doit s’accompagner d’un véritable bilan et d’une réflexion sur le modèle économique et juridique encore fragile du dispositif. Peut être les exonérations sociales et fiscales proposées au travers de cet amendement sont elles une piste,

L’article 1679 A du code général des impôts prévoit un abattement de 22 535 euros pour 2023 sur le montant annuel de la taxe sur les salaires au bénéfice des associations régies par la loi du 1 juillet 1901, des fondations reconnues d’utilité publique, des centres de lutte contre le cancer ainsi que d’autres organismes à but non lucratif. Je propose d’étendre ce dispositif aux fonds de dotation, qui sont des organismes à but non lucratif, destinés au financement de la philanthropie et du mécénat grâce à la capitalisation

Delattre justifie son amendement par la nécessité de supprimer une inégalité entre les fonds de dotation et d’autres structures, comme les associations et les fondations reconnues d’utilité publique. Toutefois, la commission est opposée au mitage de la taxe sur les salaires. Par ailleurs, elle n’a pas d’expertise particulière sur les fonds de dotation.

Patricia Schillinger. Le rapport de la mission d’information sur l’avenir de la commune et du maire en France adopté par le Sénat le 12 juillet dernier mettait en évidence une aggravation de la crise des vocations chez les élus municipaux, illustrée

Dans ce contexte, il est nécessaire de réfléchir aux moyens de faciliter l’exercice des fonctions d’élu local et, plus largement, de les rendre plus attractives afin d’attirer des candidats issus

du risque incendie : afin de faciliter la conciliation de leur activité de sapeur pompier volontaire avec leur activité professionnelle, leurs employeurs bénéficieront, à compter du 1 janvier 2024, d’une exonération des cotisations patronales. Cet amendement prévoit donc d’étendre ce dispositif aux employeurs d’élus locaux.

Il est urgent d’adopter une politique incitative l’exonération des cotisations patronales pour les entreprises qui augmenteront de 10 % les salaires de leurs salariés pendant cinq ans, dans le cadre d’un contrat d’entreprise global. Cette mesure s’appliquerait à tous les salariés gagnant jusqu’à trois fois le Smic. Cette grande mesure de pouvoir d’achat et de justice pour nos travailleurs, qui créent de la valeur et de la richesse dans notre pays, recevra – nous n’en doutons pas – votre totale approbation.

Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à supprimer l’article 10 du présent PLFSS introduit, à la hussarde, par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité à l’Assemblée nationale. Ledit article prévoit une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de dix huit mois, soit à horizon du milieu de l’année 2025, pour réformer l’assiette sociale des exploitants agricoles ultramarins. Selon le Gouvernement, « cette méthode permettrait permettrait de laisser un délai suffisant pour mener les travaux techniques et la concertation avec les organisations professionnelles agricoles, en y associant naturellement les parlementaires ultramarins l’auteur du présent amendement considère que l’alignement de l’assiette sociale des non salariés agricoles (NSA) ultramarins sur celle applicable en France hexagonale ne nécessite aucunement de passer par voie d’ordonnances. Si le Gouvernement souhaite renforcer l’acceptabilité d’une telle réforme,

l’auteur du présent amendement considère que la mise en œuvre de cette réforme majeure pour les NSA outre mer nécessite la transmission d’une expertise complète et précise permettant de mesurer les conséquences concrètes sur les prélèvements sociaux et les évolutions attendues en matière de droits pour les assurés.

Cet article habilite en effet le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures découlant de ladite réforme. Vous connaissez notre goût pour les ordonnances, en particulier le il s’agit de simplifier et de contemporanéiser les modalités de calcul et de versement des cotisations des indépendants, qui sont actuellement calculées à titre provisionnel puis régularisées lorsque les revenus définitifs sont connus. En outre, l’habilitation permettrait également au Gouvernement d’aligner l’assiette sociale des non salariés agricoles ultramarins sur celle qui s’appliquera aux indépendants de l’Hexagone, en passant d’un mode de calcul des cotisations lié à la superficie de l’exploitation à une assiette constituée des revenus professionnels. Afin de lisser les effets d’une telle transition, le Gouvernement propose d’étendre le champ des exonérations de cotisations

je tiens à rappeler qu’en juillet dernier les responsables de la filière viticole nous alertaient sur des propositions de modification de la fiscalité sur les boissons alcoolisées dans le cadre de la discussion budgétaire à venir. La question a été tranchée par Mme la Première ministre

la filière viticole est confrontée à des difficultés majeures à la suite de crises successives – crise climatique, tensions sur les marchés internationaux… En outre, cette filière est déjà soumise à une pression fiscale importante, de l’ordre de 1 milliard d’euros chaque année, sans tenir compte du foncier viticole.

La filière est engagée depuis plusieurs années en faveur d’un modèle de consommation responsable. Elle est disposée à coconstruire un projet cohérent, à partir de mesures équilibrées, pour cibler les consommations excessives sans pour autant stigmatiser une filière d’excellence. Enfin, plutôt que d’opter pour les mesures proposées, il serait plus judicieux d’investir dans des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour encourager une consommation responsable. Cela permettrait de promouvoir une approche équilibrée, tout en préservant la diversité des acteurs économiques du secteur. En conclusion, je vous encourage à reconsidérer ces amendements et à ne pas les adopter. Des Des solutions alternatives axées sur la prévention et la sensibilisation seraient plus bénéfiques tant pour l’économie que pour la santé publique. N’oublions pas que l’excédent commercial de la filière vins et spiritueux représente plus de 15 milliards d’euros. Je

et la prévention. Il faut dépasser ce clivage, travailler ensemble, trouver l’argent là où il se trouve et mettre à contribution celles et ceux qui n’ont pas d’effet positif sur nos territoires, c’est à dire les viticulteurs qui sont les plus capitalistiques et les plus internationalisés.

À force d’imposer des taxes à tout va, vous êtes en train de tuer des libertés.

les questions liées à l’avenir de cette filière. Par ailleurs, on ne peut pas admettre l’idée que l’avenir de la filière viticole repose sur une consommation maximale d’alcool

En France, le surpoids et l’obésité sont en hausse, notamment chez les jeunes. Près d’un Français sur deux est en situation de surpoids, selon l’Institut La contribution sur les boissons alcooliques comprenant des sucres ajoutés, également appelée « taxe soda », a été mise en place en 2012, dans l’objectif d’inciter les consommateurs à réduire leur consommation de sodas.

qui n’avait rien à voir avec la taxe sur les sodas, mais qui rapportait les réactions des consommateurs à une déclaration de la plus grande entreprise de sodas, une entreprise américaine – vous voyez de qui je veux parler… –, alors en pleine négociation commerciale